Madame la présidente,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 d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la désignation des membres de la mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles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

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis près de quatre ans que la délégation sénatoriale aux entreprises existe, elle sillonne la France à la rencontre des entreprises. Il ne se passe pas un déplacement de terrain sans que nous soyons interpellés sur le désavantage compétitif subi par nos entreprises lorsque la France surtranspose en droit interne certaines de ses obligations européennes. C'est en effet un vrai handicap de compétitivité qui pénalise notre économie, particulièrement notre industrie, à l'intérieur même du marché unique, par des contraintes administratives et techniques qui alourdissent les coûts et retardent la mise en oeuvre des projets.

au sujet de la surréglementation française concernant les poussières de bois, les normes européennes étant cinq fois plus basses en la matière que celles que la France a choisi de s'imposer.

le droit national allant au-delà des normes exigées par les directives ou adoptant une interprétation exigeante des règlements européens. Si tous les écarts de transposition ne sont pas illégitimes, l'impact de ces mesures nationales en termes de compétitivité est trop rarement débattu. C'est pourquoi, avec le président de la commission des affaires européennes, Jean Bizet, nous avons sollicité ce débat aujourd'hui. Le Gouvernement n'ignore pas la question. Déjà, les premiers comités interministériels pour la modernisation de l'action publique, les CIMAP, du 18 décembre 2012 et du 2 avril 2013 avaient conduit à la publication de la circulaire du 17 juillet 2013, qui prévoyait de limiter l'inflation normative, notamment de ne pas surtransposer les directives communautaires sans justification. Concernant le stock de surtranspositions, un rapport identifiant des écarts de réglementation entre la France et les autres États membres avait même été élaboré à la demande du ministre de l'économie de M. Macron, et lui avait été remis en mars 2016. Malgré tout l'intérêt de cette démarche, le gouvernement d'alors n'a malheureusement pas donné suite.

toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive, sauf justification arbitrée par le Premier ministre. Elle annonçait qu'une prochaine mission d'inspection serait chargée d'un travail d'inventaire censé aboutir en mars 2018. Bien qu'il n'ait pas été transmis au Parlement, ce travail semble avoir produit des fruits, puisque le Gouvernement vient de déposer un projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français. Sans attendre le Gouvernement, le Sénat avait pris les devants. Dès l'hiver dernier, la commission des affaires européennes et la délégation sénatoriale aux entreprises se sont mobilisées pour analyser le phénomène de surtransposition, en mesurer l'ampleur et tenter d'y remédier. Une consultation en ligne a été lancée auprès des entreprises, et notre collègue René Danesi, membre de ces deux instances, s'est vu confier le soin d'en exploiter les réponses. Sur le fondement de cas concrets, il a ainsi pu élaborer un rapport, adopté le 28 juin dernier par la délégation sénatoriale aux entreprises et par la commission des affaires européennes. Ce rapport établit une typologie des différentes situations de surtransposition et s'attache, en outre, à en identifier les motivations. Notre collègue René Danesi va donc nous présenter ses conclusions et les suites qu'il entend leur donner. Très bien

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le 28 juin dernier la commission des affaires européennes et la délégation sénatoriale aux entreprises ont adopté mon rapport d'information intitulé.

toute surtransposition susceptible de nuire aux intérêts économiques de la France, de ses filières industrielles, de ses services et de ses entreprises doit être écartée. ! Nos entreprises sont en effet pénalisées par la pratique française persistante de la surtransposition des textes européens. Il en résulte des coûts, des charges administratives injustifiées et une dissymétrie concurrentielle. À partir de cas précis étudiés dans mon rapport, j'ai dressé une typologie des surtranspositions pratiquées : extension du champ d'application de la directive, adjonction d'obligations supplémentaires, maintien d'obligations antérieures à l'harmonisation européenne et non-exploitation des facultés de dérogation ouvertes par une directive ou un règlement. En conséquence, le rapport émet vingt-six recommandations visant à prévenir de nouvelles surtranspositions ou, tout au moins, à évaluer leur impact économique. Parmi ces vingt-six recommandations, je citerai les quatre prioritaires. Premièrement, la participation active de nos administrations et des acteurs économiques aux négociations européennes pour faire prévaloir les normes et les pratiques françaises. Deuxièmement, la préparation active de la transposition, qui exige parfois une refonte en profondeur du dispositif français préexistant. Troisièmement, toute surtransposition doit être identifiée comme telle et dûment justifiée au regard de l'intérêt général qu'elle prétend protéger et qui n'aurait pas été pris en compte dans le texte européen. En outre, l'impact d'une surtransposition sur les entreprises doit faire l'objet d'une évaluation économique documentée. Quatrièmement, j'appelle particulièrement votre attention sur les insuffisances de la pratique des transpositions par voie d'ordonnance. Le Parlement doit être en mesure de les examiner pour corriger, s'il y a lieu, les écarts de transposition défavorables à nos entreprises. Le Gouvernement est également conscient du problème, puisqu'il a déposé sur le bureau du Sénat un projet de loi visant à supprimer vingt-sept surtranspositions existantes dans le droit français. Ce projet de loi a été examiné hier par la commission spéciale que j'ai l'honneur de présider. Il est inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée mardi prochain. Il s'agit, à mon sens, d'une première étape. Le Gouvernement doit poursuivre l'examen des surtranspositions identifiées, en particulier par une mission inter-inspections, et en supprimer l'essentiel dans son domaine réglementaire.

secrétaire d'État, que nous attendons avec impatience le rapport du Gouvernement sur les surtranspositions prévues par la loi pour un État au service d'une société de confiance. Mais nous ne nous contenterons pas d'attendre. La présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, le président de la commission des affaires européennes et moi-même venons de déposer une proposition de résolution invitant le Gouvernement à revenir sans tarder sur des surtranspositions réglementaires existantes particulièrement pénalisantes pour les entreprises. Enfin, le Sénat traduira sa volonté de voir traiter le stock existant de surtranspositions législatives

monsieur le président de la commission des affaires européennes, madame la présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de débattre de ce sujet avec vous aujourd'hui dans le cadre de votre semaine de contrôle. La dé-surtransposition de notre droit a un impact très concret sur nos entreprises et sur la vie quotidienne des Français. Le Président de la République et le Premier ministre, vous le savez, ont pris des engagements politiques forts pour sortir d'une logique qui consistait à complexifier le droit européen sans apporter de réels bénéfices aux entreprises et aux Français. Je tiens donc à remercier la commission des affaires européennes et la délégation sénatoriale aux entreprises d'avoir demandé ce débat spécifique. Vous vous inscrivez dans une séquence particulièrement riche sur le sujet.

Comme vous le savez, le Président de la République et le Premier ministre ont fait du sujet des surtranspositions une priorité politique. Pendant trop longtemps, nous avons eu tendance à faire du droit européen une base de travail que nous pouvions raffiner sans limites, sans voir les contraintes que cela créait pour les entreprises françaises. Il y avait au moins trois méthodes de surtransposition. La première consistait à laisser subsister, par inertie ou dans un souhait de fidélité louable à nos traditions juridiques, des règles préexistantes, parfois anciennes, et, en règle générale, plus contraignantes que celles promues par le droit européen. La deuxième méthode consistait à aller délibérément au-delà du standard fixé par la norme européenne, qui est le plus souvent un standard minimum, et d'inscrire directement en droit français une nouvelle règle, parfois plus sophistiquée, souvent plus contraignante. La troisième méthode consistait à ne pas faire usage d'options prévues par le législateur européen permettant un régime simplifié dans certains cas ou pour certaines catégories d'acteurs économiques, en particulier les petites entreprises. entreprises. Ces manières de faire ont abouti à complexifier le droit en créant de nouvelles contraintes et elles ont entraîné un manque de lisibilité sans apporter de réelles garanties nouvelles, ni aux entreprises françaises, qui se voyaient concurrencées par des entreprises de pays voisins appliquant un droit plus simple ou plus souple, ni à nos concitoyens, dans la mesure où la complexité des normes l'emportait souvent sur les protections offertes au plan national. C'est pour cette raison que le Gouvernement

Plus nous aurons un droit français surtransposé, plus il sera complexe pour nos entreprises de s'implanter dans les pays européens et plus il sera difficile pour une entreprise étrangère de s'implanter en France. L'Europe doit redevenir un terrain d'opportunités économiques pour nos entreprises, et non une contrainte subie. Le Premier ministre a fixé deux règles pour limiter les transpositions de directives. La première est l'arrêt de toute nouvelle surtransposition qui ne refléterait pas un choix politique assumé pour défendre les intérêts de nos entreprises ou pour protéger les Français la seconde est la mise en place d'une procédure spécifique d'autorisation du Premier ministre. Pour accompagner ces nouvelles règles, nous avons appliqué un principe d'évaluation systématique lors des transpositions du droit européen. Nous avons ainsi procédé à une évaluation du stock des surtranspositions existantes et mené une mission inter-inspections afin de corriger celles qui devaient l'être. Cela a permis d'identifier des mesures de dé-surtransposition, qui sont portées dans les différents véhicules présentés par le Gouvernement depuis le début du quinquennat,

Cela signifie-t-il la fin de toute surtransposition ? Non, car il peut y avoir de très bonnes raisons de surtransposer : pour protéger les consommateurs ou garantir des conditions de sécurité en matière environnementale ou sanitaire. Nous assumons certains standards plus protecteurs qui vont au-delà des normes européennes minimales, car ils répondent à nos préférences collectives pour mieux protéger les entreprises et les citoyens. Nous ne proposons donc pas une dé-surtransposition sauvage qui abandonnerait nos intérêts économiques, notre intérêt public et notre souveraineté juridique. C'est une affaire d'équilibre et d'appréciation au cas par cas. Le Gouvernement ne soutient pas l'idée d'une Europe qui signifierait systématiquement un nivellement par le bas. C'est pourquoi nous continuerons à nous battre pour des standards européens ambitieux dans tous les domaines.

qui est en cours d'examen par votre assemblée. Cette politique d'harmonisation de notre droit au niveau européen, nous la menons avant tout pour simplifier la vie des entreprises. Si je devais citer un exemple, ce serait l'allégement des obligations comptables pour les moyennes entreprises.

Le premier concerne les seuils de certification légale des comptes, que nous relevons au niveau des seuils de référence proposés par le droit européen. Nous avons soumis cette surtransposition à une étude d'impact approfondie et rigoureuse, qui a démontré que le coût engendré par cette obligation s'élevait à 5 500 euros en moyenne par an pour les entreprises situées en dessous des seuils et qu'il n'était pas associé à un bénéfice quantifiable en matière de fiabilité des états comptables et fiscaux.

le combat est important pour obtenir des activités complémentaires dans le cadre du Brexit. Tels sont la logique que nous voulons mettre en place, les engagements politiques que nous avons pris et notre méthode. Je vous propose maintenant d'entrer dans le détail en répondant à vos questions pendant ce

Certes, il y a une inflation législative et la loi est souvent bavarde, créant une complexité pour les citoyens, les usagers des services publics ou encore les entreprises. De réforme en réforme, en lieu et place de l'efficacité se profile une véritable insécurité juridique- nous avons eu l'occasion de le rappeler maintes fois dans cette enceinte. de la surtransposition est à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit d'aller au-delà des directives de libéralisation ou d'ouverture à la concurrence de nos services publics, je le dis, chers collègues, peu de voix s'élèvent dans cet hémicycle. Par contre, il y a une forme d'unanimité de la droite sénatoriale et de la droite gouvernementale pour s'opposer à toute règle nationale plus protectrice que le droit européen. Ainsi, le rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises déplore que la surtransposition rende applicable au plan national le standard que la France n'a pu imposer au niveau européen en matière de sécurité et de santé au travail, de préservation de l'environnement et de la biodiversité, de protection des consommateurs ou encore de transparence de l'action publique. Nous pensons au contraire que c'est une bonne chose, d'autant que nous parlons de directives qui laissent une marge de souveraineté aux États membres, et non de règlements européens.

Aujourd'hui, une législation plus protectrice des citoyens et de l'environnement ou un renforcement de la sécurité alimentaire sont décriés comme entraînant des coûts insupportables pour nos entreprises, alors que ces mesures devraient être saluées. Ma question comment justifiez-vous que seul le supposé coût économique soit pris en compte pour faire la part entre une bonne et une mauvaise surtransposition, alors que ce sont la santé des travailleurs, la protection de l'environnement ou encore la sécurité des consommateurs qui sont en jeu ? La parole est à Mme la secrétaire

On dit que c'est un mal français. La surtransposition des normes est en tout cas un vrai serpent de mer. Enquêtes, débats et rapports se succèdent depuis des années, avec des conclusions souvent tranchées : rigidité pour certains, protection pour d'autres

Et si la vérité était plus nuancée ? Ce sont les gouvernements successifs et les législateurs que nous sommes qui font la loi. Nous sommes donc coresponsables de la situation que nous dénonçons. D'abord, il y a ces pressions de plus en plus nombreuses, fréquentes et organisées. Ces groupes ont une force de frappe énorme. Résultat : au travers des voix des parlementaires, ce sont quelquefois les lobbys qui s'opposent. S'ils ont tant de prise sur le Parlement, interrogeons-nous sur les causes : la course à légiférer limite le temps de la réflexion et surtout l'analyse des impacts de nos décisions. Sur le terrain, les citoyens, les élus, les chefs d'entreprise nous interpellent sur notre décalage avec leur réalité. Derrière le sujet de la surtransposition des normes se posent d'autres enjeux : nos insuffisances réelles- pédagogie, concertation, simplification, impacts ... Autant d'étapes minimisées qui conduisent à pénaliser nos entreprises, à immobiliser des projets structurants. Notre collègue René Danesi pointe l'incapacité de la France à participer au processus de discussion des projets européens. C'est un reflet de notre incapacité au niveau national. Les positions sont clivées dès le départ, et le rythme imposé est un déni du débat démocratique. Cela conduit à des postures politiciennes au sein du Parlement et,, à des interprétations de nos administrations, qui jonglent souvent avec les doctrines de plusieurs ministres. Au-delà de l'élimination de surtranspositions, qui aura pour effet de récuser des intentions parfois fondées de protection sociale et environnementale, il faudrait élaborer une méthode.

travaillé à mettre plus de concertation dans nos, plus de réflexion dans la façon de conduire nos réformes et à mieux prendre en

Madame la secrétaire d'État, beaucoup de transporteurs locaux ont orienté une partie de leur activité vers l'utilisation de solutions multimodales rail-route-eau pour desservir les ports du Sud et ceux de la mer du Nord. Cette solution optimise les plans de chargement des industriels et les volumes transportés par voyage, représentant une augmentation de 15 %. Elle permet aussi de réduire proportionnellement le nombre de mouvements de camions, en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, transposée en 1997 dans le code de la route, détermine des normes en matière de poids et de dimension des véhicules. Elle autorise le transport international de marchandises par des ensembles de poids maximal de 44 tonnes uniquement dans des cas de transport intermodal. Force est de constater que beaucoup de transporteurs étrangers, défiant ces règles de transport modal, profitent d'une lacune de transposition de la directive européenne pour transporter sur nos routes des conteneurs surchargés. En contournant En contournant la loi, ils créent de fait une concurrence déloyale, susceptible de mettre en péril le modèle économique multimodal. Si l'exercice du contrôle sur le volet spécifique du passage du passage de frontière par des ensembles routiers transportant des conteneurs en surcharge est possible, il n'existe pas de transposition des sanctions prévues par le droit européen dans le droit français.

Nous souhaitons plus de transparence sur les modalités d'application et de contrôle de ces règles pour les transporteurs, notamment internationaux. Vous avez évoqué des situations où la concurrence est mise en cause, parce que des transporteurs internationaux ne respectent pas les règles.

est source de bien des difficultés pour nos entreprises. D'ailleurs, nous sommes tous ici régulièrement interpellés à ce sujet dans nos départements. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, mais aussi les agriculteurs et les industriels, tous souffrent de la distorsion de concurrence avec nos voisins européens que ce phénomène implique. En tant que frontalier, j'en parle en connaissance de cause. Sur des sujets cruciaux, comme l'environnement, pour ne citer que cet exemple, la France impose à ses entreprises des objectifs et des normes plus contraignants que ceux auxquels sont soumises les autres entreprises européennes. Cette distorsion est bien évidemment préjudiciable à l'attractivité économique de notre pays. Cela est particulièrement prégnant dans le contexte du Brexit. En effet, de nombreuses entreprises de toute nature, actuellement implantées au Royaume-Uni, vont être amenées à localiser ou relocaliser leur activité sur le continent. L'implantation d'acteurs économiques depuis le Royaume-Uni devrait constituer une opportunité de développement plus que bienvenue pour certains de nos territoires. Encore faut-il que ces entreprises fassent le choix de la France ! Pour cela, notre réglementation ne doit pas être plus contraignante que celle de nos voisins, à plus forte raison quand elle est issue de textes communautaires. Dans le projet de loi visant à supprimer certaines surtranspositions, qui est actuellement examiné par le Sénat, une mesure en particulier est tournée vers l'attractivité de la place financière de Paris, avec l'objectif d'attirer vers notre capitale les firmes de la City. C'est une ambition légitime, mais la finance ne doit pas nous faire oublier les autres domaines d'activité économique dans lesquels nous devons renforcer notre attractivité.

Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement a engagé un plan ambitieux en faveur de l'attractivité de la place financière française, car nous avons la conviction que le secteur financier- et pas seulement celui-là, puisque, vous le savez, une mission a été confiée à Ross McInnes sur la dimension industrielle -est un atout pour nos entreprises et pour l'emploi.

qui pouvaient être pris en compte dans sa décision ; j'y reviendrai. Dans le cadre des mesures annoncées par le Premier ministre en juillet 2017 puis en juillet 2018, la simplification réglementaire et la dé-surtransposition du droit financier ont eu toute leur place, aux côtés de mesures visant à améliorer la structure de coûts des entreprises financières. Je veux en citer trois exemples : la suppression de l'obligation faite aux chambres de compensation d'obtenir un agrément d'établissement de crédit, la limitation des surtranspositions applicables aux sociétés cotées et l'élargissement de l'accès au système de paiement et de règlement-livraison. Il est clair aujourd'hui que l'un des sujets qui demeurent est celui de l'écart de compétitivité-coût,

La parole est à M. Jean-Pierre Decool. Le débat qui nous occupe aujourd'hui interroge tout à la fois les relations entre le législateur national et le législateur européen, ainsi que la stratégie d'influence de la France

Nous ne devons pas avoir comme seule boussole l'alignement systématique sur la norme européenne. Nous devons veiller, comme le propose notre collègue Danesi, à évaluer les surtranspositions préjudiciables à nos entreprises. travail fait, nous devons encore arbitrer entre le préjudice subi et l'intérêt général poursuivi par le législateur. Deuxièmement, ces surtranspositions marquent souvent l'échec de l'influence française au sein du processus décisionnel européen. Nous sommes trop peu présents dans les consultations et les négociations qui précèdent l'adoption des actes européens ou encore au sein des comités techniques européens. Notre modèle d'influence, fondé sur la bicéphalie entre la représentation permanente et le secrétariat général des affaires européennes, est souvent critiqué pour sa lourdeur. De même, le monde économique n'est pas suffisamment intégré aux négociations en amont du processus de transposition. Ma question, madame la secrétaire d'État, porte sur la stratégie d'influence de la France au sein des institutions.

européenne ambitieuse dans les propos et sa politique d'influence, parfois moins efficace que celle d'autres États qui savaient diablement bien tirer leur épingle du jeu dans les négociations multilatérales.

Nous avons noué des contacts au niveau diplomatique avec les parlementaires européens, avec les représentations des États, avec les parties prenantes du débat européen. Nous travaillons le plus en amont possible pour faire valoir des objectifs et les concilier avec les manières de voir d'autres pays, parce qu'il s'agit bien de négociations et de prise en compte de tous les points de vue. Il faut aussi accepter de se décentrer quelque peu. C'est la démarche que nous adoptons, par exemple, sur la fiscalité du numérique, pour laquelle nous prenons le temps d'essayer de construire une position commune. Vous savez comme moi combien c'est difficile. En ce qui concerne les entreprises, il nous paraît essentiel de les consulter, mais de le faire avec les plus fortes garanties de transparence et d'objectivité, car nous savons que le projet européen souffre aussi de soupçons de capture d'intérêts économiques par nos concitoyens. Je pense que vous y êtes sensible, puisque vous avez affirmé que la surtransposition n'était pas nécessairement négative. Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite pouvoir entendre le point de vue de tous les acteurs- entreprises, ONG, experts issus du monde académique et société civile

savoir le Conseil national d'évaluation des normes. J'entends également parler de la création d'une instance chargée d'interpeller ces mêmes pouvoirs publics sur les lois qui, cette fois, auraient un impact négatif sur les entreprises. Comment en sommes-nous arrivés là ? Madame la secrétaire d'État, les surtranspositions sont, à mon sens, le résultat d'un État qui peine à faire appliquer ses lois et qui ne cesse d'en créer de nouvelles, en espérant que l'une d'elles soit enfin entendue. De cette boulimie législative résultent des failles dans les relations entre les équipes chargées des négociations européennes et celles qui ont la charge de la transposition, mais aussi des lacunes dans les études d'impact. Bref, la machine s'est emballée, et plus personne ne s'y retrouve. que la solution réside dans la capacité des gouvernements à faire appliquer les lois existantes, notamment en donnant aux douanes les moyens de faire leur travail ? Pour gagner en lisibilité, ne pensez-vous pas que la solution réside peut-être dans des lois moins nombreuses, mais appliquées ? Lorsque l'on sait que, faute de décrets d'application, un tiers des lois n'est pas mis en oeuvre, ne pensez-vous pas que, pour faire cesser cet emballement législatif et ces surtranspositions nuisibles, la parution des décrets d'application doit être plus rapide ? Quant aux lois « d'affichage » inapplicables, qui ne font que nourrir les revues juridiques, les sénateurs et, je l'espère, les députés sont assez responsables pour y mettre fin. La parole est à Mme la secrétaire

» Je crois percevoir dans vos propos l'idée que les surtranspositions et l'affluence de normes ne sont pas de nature à améliorer la réalité de notre action publique. Je partage votre souhait de simplifier nos règles pour faire progresser le niveau de protection de nos concitoyens, pour les rendre lisibles et donc applicables. À ce titre, plusieurs principes me paraissent devoir être observés : le respect

Tous nos projets de loi sectoriels doivent comporter un volet de simplification. Nous savons collectivement que c'est difficile, puisque nous avons tous envie d'influencer la trajectoire de la décision publique- c'est peut-être un péché mignon que nous partageons ... Sachez néanmoins que

Nous avons adopté à l'unanimité le texte visant à confier à des cabinets indépendants les études d'impact des textes discutés. La Questure du Sénat vient d'ailleurs de lancer un appel d'offres à ce sujet. Les mêmes questions se posent dans les mêmes termes au niveau européen

Dans son avis sur le projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français, le Conseil d'État « regrette que l'étude d'impact, [ ...], n'indique pas, [ ...], les motifs [ ...] pour lesquels les dispositions [ ...] avaient été en leur temps introduites en droit interne et le contexte dans lequel ces choix de transposition ont été faits

Ces remarques pourraient tout autant s'appliquer au processus de transposition des directives dans le droit national. Madame la secrétaire d'État, pour la clarté du débat parlementaire, une plus grande efficacité des transpositions et la limitation au strict nécessaire, dûment justifié, des surtranspositions, envisagez-vous la mise en oeuvre d'études d'impact des directives transposées et, si oui, suivant quelles modalités et quel calendrier de mise en oeuvre ? La parole est à Mme la secrétaire Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous le savez comme moi, les études d'impact des projets de loi et des actes réglementaires prévoient systématiquement une analyse du texte au regard du droit européen.

En Europe, les populismes montent. La démocratie n'est plus considérée par beaucoup d'Européens comme « le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres », comme le disait Winston Churchill. La vie au quotidien des citoyens européens et des entreprises est davantage régie par le droit de source européenne que par les droits nationaux. Comme un moyen parmi d'autres, la publication d'études d'impact véritablement indépendantes relatives aux transpositions et à l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques européennes permettrait de donner plus de sens politique et démocratique à la construction européenne.

Nous regrettons cependant, madame la secrétaire d'État, que le Parlement ne soit pas davantage associé au processus de lutte contre les excès de transposition des directives européennes. Le Sénat a pourtant été à l'origine de nombreux rapports mettant en évidence

de plus long terme et de plus grande ampleur. Aujourd'hui, les parlementaires saisis des projets de loi portant transposition de directives européennes disposent en général de peu de temps pour les examiner en détail, détail, d'autant qu'il s'agit souvent de mesures particulièrement techniques. Repérer et surtout évaluer les différentes surtranspositions peut donc être, dans ce contexte, une tâche ardue. revanche, les Parlements nationaux étaient associés en amont de la négociation des directives elles-mêmes, le travail sur la transposition de ces textes pourrait s'effectuer de manière à la fois plus approfondie et plus apaisée. Ainsi, madame la secrétaire pouvez-vous nous assurer que le Parlement aura toute sa place dans le processus de lutte contre les surtranspositions présentes et, surtout, de prévention des surtranspositions futures ? La parole est à Mme la secrétaire

des enjeux liés à la réglementation européenne que nous progresserons dans notre effort d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens et de nos entreprises. C'est pour cette raison que le Gouvernement est à l'écoute des préoccupations des parlementaires et qu'il leur transmet des éléments d'information sur les négociations en cours. Comme vous le savez, ces négociations peuvent s'étirer et ne sont pas toujours

Je ne peux donc que vous assurer de notre volonté d'approfondir cette démarche, dès lors qu'elle est de nature à favoriser une meilleure compétitivité de la France, une meilleure lisibilité de notre droit et une capacité à augmenter collectivement le niveau de protection de nos concitoyens.

Pour conforter la position de la France en tant que mondial du tourisme et atteindre l'objectif de 100 millions de touristes internationaux en 2020, le Gouvernement a fait un certain nombre d'annonces pour développer le secteur touristique. qu'élue d'un territoire de montagne, les Hautes-Alpes, je ne peux que m'en réjouir, puisque, avec 53,8 millions de journées-skieurs, les massifs français sont la deuxième destination mondiale pour le ski, derrière l'Autriche. Les stations représentent 120 000 emplois induits et toute une économie construite autour des remontées mécaniques. C'est pourquoi je veux appeler votre attention sur les seuils applicables aux aménagements des domaines skiables aux termes de l'article R. 122-2 du code l'environnement. Contrairement à nos voisins des pays de l'arc alpin, ces seuils ont été fixés à un niveau très bas, entraînant un examen systématique au cas par cas, avec, souvent, l'obligation d'une étude d'impact pour des aménagements dont la taille et les effets supposés sur l'environnement ne la justifient pas. Pis, lorsqu'il s'agit du remplacement d'un appareil de remontée mécanique, une étude est aussi nécessaire, alors que l'on se trouve exactement dans le même périmètre.

réalisation d'une étude d'impact nécessite un délai minimal de douze mois pour l'observation de la faune et de la flore et entraîne une enquête publique, donc des délais supplémentaires. supplémentaires. Afin de mettre fin aux surtranspositions françaises qui pénalisent l'économie montagnarde, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m'indiquer si,

qui, par volonté politique, opte pour des dispositions plus restrictives ou des objectifs plus contraignants que la directive encadrant le domaine d'intervention, mais conformes à l'éthique de responsabilité et aux attentes des citoyens. Je pense, par exemple, à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en France à 23 % en 2020 et à 32 % en 2030, alors que la directive du 23 avril 2009 ne fixait qu'un objectif minimal de 20 % en 2020. Oui, c'est un choix politique, qui sous-tend d'ailleurs la montée en puissance de secteurs économiques qui ont besoin de ce type de signal pour prospérer ! Voilà un exemple de surtransposition bienvenue pour notre économie ! Le mécanisme n'est donc pas toujours en défaveur de nos entreprises. Autre exemple : les pesticides. Je suis d'autant plus concerné par ce sujet que le Gouvernement vient de prendre la décision unilatérale d'interdire la substance active métam-sodium à la suite de l'intoxication de plusieurs dizaines de personnes provoquée par la pulvérisation de ce produit dans mon département de Maine-et-Loire, pour préparer la culture de la mâche. Je partage l'idée d'une nécessaire simplification du droit là où c'est possible. Mais attention à ne pas rogner trop hâtivement notre droit de l'environnement ou de la consommation sur l'autel de la concurrence libre et non faussée ! D'où ma question, madame la secrétaire d'État : le rapport de notre collègue propose par exemple dans sa recommandation première « de mieux associer le monde économique aux négociations sur les projets d'actes législatifs européens en amont de la transposition ». Mais il semble ici que l'on oublie les consommateurs et les usagers. Une solution équilibrée proposée par le Conseil d'État en 2016 semble plus plus adaptée, à savoir la création « d'un conseil unique d'évaluation des normes doté de trois collèges représentant les usagers, les collectivités territoriales et les entreprises ». Que pensez-vous de cette approche tripartite en matière de surtransposition ? La parole est

Nous assumons ces standards plus protecteurs qui vont au-delà des normes européennes minimales, car ils répondent à nos préférences collectives pour mieux protéger les entreprises et les citoyens. Nous ne proposons donc pas, comme je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, une dé-surtransposition sauvage qui abandonnerait nos intérêts économiques, notre intérêt public ou notre souveraineté juridique.

La parole est à M. Daniel Gremillet. Le constat est posé : la compétitivité de notre économie se trouve trop souvent entravée par des contraintes purement nationales, qui viennent s'ajouter aux objectifs fixés par les directives européennes. Pourtant, l'impact de ces mesures nationales en termes de compétitivité, de charges administratives et de garanties données aux citoyens, par rapport à nos voisins européens, n'est quasiment jamais débattu.

René Danesi. L'enjeu est avant tout d'ordre économique : en imposant à ses entreprises des normes plus contraignantes que celles qui sont en vigueur dans les autres États membres, quel que soit le secteur concerné, la France se met en situation de fragilité. Et pour quel résultat ? Cette pratique française interroge et peut être comparée à la situation qui prévaut en Allemagne, où, selon un principe simple, toute surtransposition est interdite, sauf si elle est favorable aux entreprises nationales et dûment justifiée. Plus largement, je souhaiterais que la France soit plus stratège et ambitieuse à l'égard des entreprises et des acteurs économiques français. Ces travaux ont révélé que le droit français comporte un certain nombre d'obligations de publicité qui conduisent à informer la concurrence de projets innovants ou à leur donner accès à des informations confidentielles.

De manière surprenante, la surtransposition du droit européen en France empêche le développement des entreprises de production d'énergies renouvelables. Le cas de la production d'électricité issue de la petite hydroélectricité est à cet égard très révélateur et alarmant. En effet, quand la directive européenne sur les continuités écologiques, dite DCE, est transposée en France, on surtranspose ! Plus précisément, l'administration surtranspose sans vergogne Certes, l'autorité administrative française dispose des moyens d'établir les prescriptions nécessaires au respect de la gestion équilibrée des cours d'eau ; toutefois, surajoute des contraintes dans l'utilisation de nos cours d'eau, elle surdécline le concept de continuité écologique à travers une kyrielle de lois et de règlements, qui s'ajoutent les uns aux autres et vont, en ce sens, au-delà de la simple transposition du concept issu de la DCE.

Et je ne parle pas de l'arrêté de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, qui impose toutes sortes de mesures au titre de la préservation de la continuité écologique sur les cours d'eau non classés classés ni du projet de décret relatif à la continuité écologique, qui risque d'en rajouter une couche ! Le préjudice est d'ampleur pour le développement des énergies renouvelables : sont perdus de vue les principes de gestion équilibrée et de conciliation des usages, pourtant inscrits dans le code de l'environnement. Et la surtransposition crée une instabilité économique et juridique, en précarisant lesdits ouvrages hydroélectriques et leur exploitation ! On oublie qu'une autre directive européenne sur les énergies renouvelables et la loi du 17 juillet 2015 sur la transition énergétique prônent le développement des énergies renouvelables,

des objectifs environnementaux avec des objectifs d'accès à l'eau. Vous savez que des pompages trop importants peuvent aussi déstabiliser des zones hydriques. Ce ne sont pas simplement

dans cet objectif de respect de l'environnement et de mixité des usages. Soyez assuré que, s'agissant des énergies renouvelables, nous sommes très fortement engagés dans ce

Parmi ces entreprises, il y a bien évidemment les entreprises agricoles, auxquelles je souhaite consacrer ma question. Les élevages français sont pénalisés par rapport à leurs concurrents européens du fait de la surtransposition de la directive européenne sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés, En droit français, pour les élevages de porcs et de volailles, les seuils imposant à un projet d'élevage de réaliser une étude d'impact sur l'environnement, préalable à une demande d'autorisation d'exploiter, sont plus contraignants que les seuils fixés par la directive directive EIE. Un projet d'élevage français est soumis à cette obligation tandis qu'un projet de même nature dans un autre État membre en sera dispensé. Cette surtransposition est pénalisante pour les élevages de porcs et de volailles dans la mesure où où la réalisation d'une étude d'impact est longue et coûteuse. Cela ne fait que s'ajouter à la longue liste des contraintes administratives qu'on leur impose. Cette surtransposition est de niveau réglementaire et non législatif, elle ne peut donc être directement supprimée dans le cadre d'un projet de loi comme celui qui, hasard du calendrier, vient en discussion la semaine prochaine- et qui, au passage, manque nettement d'ambition. Ma question est donc simple : quelles actions le Gouvernement prévoit-il de mettre en oeuvre pour lutter contre les surtranspositions d'origine réglementaire, notamment la surtransposition de la directive EIE, qui pénalise les élevages français de porcs et de volailles ? Excellente question Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, conformément à une promesse du Président de la République, le Gouvernement a lancé l'année dernière des états généraux de l'alimentation. Ceux-ci avaient pour objectif de mieux rémunérer les agriculteurs tout en augmentant la qualité de l'offre française. La concurrence européenne, vous l'avez souligné, ne doit donc pas être synonyme de moins-disant réglementaire, mais nous ne devons pas être naïfs, et l'élevage est un secteur soumis à une concurrence internationale féroce. Des mesures de simplification, de dé-surtransposition, ont été adoptées ces dernières années, notamment s'agissant des installations classées pour la protection de l'environnement. Il me semble- je l'entends dans votre propos -que l'on peut aller plus loin.

Nous constatons ainsi sur nos routes des transporteurs européens qui font des opérations de cabotage sans ces contraintes. Ces lois ou règlements français, qui vont au-delà des exigences fixées par l'Europe, pourraient se défendre si nous n'étions pas un pays ouvert au libre-échange et à la concurrence internationale. Ce n'est pas l'orientation qui a été prise. Nous avons fait le choix de défendre notre pouvoir d'achat en optant pour la libre concurrence. Je le respecte. Les entreprises françaises doivent donc être compétitives pour pouvoir vendre leurs produits. Or elles ont un coût horaire de travail qui est quatre fois supérieur à celui de pays voisins comme la Pologne. Si, en plus de la question du social, que nous n'avons toujours pas réglée, nous continuons de produire des lois ou des règlements uniquement français, nous diminuons encore nos chances de voir se développer ou se transmettre nos entreprises de petite et moyenne taille, de voir les plus grosses, qui sont internationales, optimiser leurs résultats par rapport aux pays les moins taxés. Nous risquons également d'avoir à supporter les pertes de recettes fiscales des GAFA.

la transposition des directives en droit français et les mesures d'application des règlements européens. En début d'année, la conférence des présidents l'a chargée, à titre expérimental, d'une mission de suivi des transpositions. Elle examine les projets et propositions de loi pour en évaluer sous ce regard la qualité de la transposition proposée et attirer l'attention de la commission saisie au fond sur les écarts de transposition. Elle a ainsi été conduite à exercer cette mission de vigilance dans le cadre de trois textes adoptés au cours des derniers mois : en matière de protection des secrets d'affaires ; en matière d'encadrement des services de paiement en matière de mise en oeuvre du règlement général de protection des données à caractère personnel. Le projet de loi PACTE sera une nouvelle occasion d'exercer cette mission, qui est, faut-il le préciser, en parfaite cohérence avec le rôle qui incombe à la commission des affaires européenne du Sénat dans le cadre de l'élaboration des textes européens. Les propositions de résolution qu'elle adopte pour attirer l'attention du Gouvernement sur les enjeux attachés aux travaux d'harmonisation en cours au niveau européen et les avis politiques qu'elle adresse à la Commission et au Parlement mettent en particulier l'accent sur la définition du périmètre qu'il est proposé d'harmoniser, sur la pertinence de la portée de l'harmonisation proposée et sur l'adaptation du traitement réservé aux préoccupations françaises en matière de protection des consommateurs, de lutte contre la fraude, de protection raisonnée et raisonnable de l'environnement ou encore de santé publique. Nous nous efforçons de suivre les travaux européens, de mesurer les conséquences potentielles des mesures proposées pour nos opérateurs économiques. Le droit européen ne doit pas être appréhendé comme un recul du cadre national, mais comme l'occasion de promouvoir notre modèle au niveau européen, tout en permettant à nos entreprises de ne pas être pénalisées par des règles nationales que ne supportent pas leurs concurrentes, en termes de charges administratives, de coûts et de contraintes de production.

Des améliorations méthodologiques doivent être apportées sans tarder à la participation française au processus d'élaboration du droit européen comme à la procédure de transposition du droit européen en droit français.

du Conseil d'État dans son étude de 2015. Toute mesure de surtransposition doit être dûment identifiée et justifiée. Il y a là véritablement un nouvel état d'esprit à insuffler, responsable et positif. Nous comptons sur le Gouvernement pour jouer pleinement le rôle qui lui incombe en la matière, pour appuyer les observations du Parlement et le tenir beaucoup mieux informé des évolutions des négociations au niveau européen, pour lui fournir les éléments dont il a besoin pour évaluer les conséquences des surtranspositions proposées. La prise de conscience de l'importance d'une telle approche constitue une première étape positive. Il convient qu'elle soit généralisée et mise en oeuvre dans la durée. Nous sommes sensibles à la détermination affichée en la matière par le Gouvernement.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement bénéficiera de la même durée pour lui

avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes remerciements au président Alain Milon pour la confiance témoignée au moment du lancement du groupe de travail sur l'accompagnement du handicap et à mes collègues de la commission des affaires sociales pour leur engagement au cours de ces dix mois de travail.

des affaires sociales. Dans ce rapport, j'ai suggéré quarante propositions. Je ne peux pas les présenter toutes à cette tribune, mais je vous ferai part de deux grandes orientations qui sont à mes yeux particulièrement importantes. La première a trait à la simplification de l'offre médico-sociale destinée aux personnes handicapées. Alors que nous entamerons, la semaine prochaine, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce sujet ne me paraît plus pouvoir souffrir de report. Les acteurs de l'accompagnement et les personnes handicapées sont unanimes dans leur souhait de voir s'améliorer la situation pour éviter des parcours inutilement complexes, des contraintes administratives et financières empilées qui limitent l'épanouissement des personnes et leur intégration dans la cité. Cette complexité, mes chers collègues, est le fruit de notre histoire. On pourrait, à bon droit, me répondre que, depuis la loi du 11 février 2005, ce principe simple et distinct se nomme « société inclusive désignant de ces deux mots forts l'ambition de faire à toute personne handicapée une place dans la société qui tient compte de sa situation particulière. Mais c'est à mon sens confondre la destination et la traversée. Si le cap est partagé, les difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans leur vie quotidienne, dans leur accompagnement à domicile ou en établissement, n'ont pas connu, depuis 2005, d'atténuation particulière. Pis, la complexité de leur parcours s'est aggravée. Le constat revient fréquemment : les parcours ne se mesurent pas à l'aune des personnes, mais à celles des structures. Voilà plusieurs années que les gouvernements successifs ont pris conscience des écueils d'un modèle d'accompagnement qui se définit essentiellement par l'offre. Encore aujourd'hui, le principal déterminant d'une couverture territoriale, suffisamment étoffée, reste le nombre de places. Cet indicateur réduit l'accompagnement à la qualification d'un établissement ou d'un service unique et n'en traduit que très imparfaitement la pertinence. Le pilotage par le nombre de places entretient par ailleurs un tropisme de la structure et maintient d'importants cloisonnements entre acteurs de l'accompagnement, là où l'on souhaite, au contraire, introduire plus de fluidité et de porosité. Pour ce qui regarde le travail des personnes handicapées, je propose que l'ensemble des acteurs publics chargés de leur insertion et de leur maintien dans l'emploi soient réunis dans un seul et même service public de l'emploi. Pour ce qui relève de l'accompagnement médico-social, il me paraît certes indispensable que les gestionnaires d'établissements et de services disposent d'une certaine liberté d'administration pour proposer des parcours plus modulaires. Toutefois, cette liberté doit être précisée au travers des instruments juridiques par lesquels ils contractualisent avec leur autorité tarifaire. Pour rompre avec les travers d'une offre médico-sociale excessivement descendante, qui privilégie l'injonction statistique des bureaux centraux par rapport aux besoins réels du terrain, il est évident que la main doit être laissée à ceux qui accompagnent directement la personne. Mais veillons à ce que ces parcours, construits au plus près des personnes concernées, ne les enferment pas dans de longs dispositifs intégrés, où les ruptures seraient certes moins fréquentes, mais où l'accompagnement s'éloignerait tout autant des attentes exprimées ... Cela m'amène au second point que je souhaitais soulever. Le grand défaut de notre modèle réside dans l'écoute très insuffisante des besoins des personnes handicapées, qui devraient seuls guider la réponse que nous devons leur apporter. Or, en la matière, les progrès sont beaucoup trop timides. les MDPH, qui sont nos acteurs de première ligne, ne sont pas habilitées à porter un diagnostic circonstancié et territorialisé des besoins exprimés dans leur département. Elles ne sont là que pour rendre compte de la somme des besoins individuels qu'elles recueillent et qu'elles essaient de faire correspondre à une offre territoriale sur laquelle elles n'ont pas la moindre prise.

Il s'agirait d'une structure territoriale dédiée, intervenant à l'échelon le plus pertinent, celui du bassin de vie, et réunissant l'ensemble des acteurs concernés par le parcours de vie d'une personne handicapée. Trois missions lui seraient assignées. Premièrement, après un recensement des besoins, la plateforme territoriale du handicap livrerait le produit de ses réflexions aux instances décisionnaires locales et nationales qui, chargées du redéploiement de l'offre, disposeraient alors d'une base quantitative et, surtout, qualitative suffisamment dense et circonstanciée pour prendre les décisions d'autorisation et d'implantation. Deuxièmement, la PTH jouerait également un rôle d'animation et de coordination auprès de tous les acteurs du handicap intervenant sur le bassin de vie. Troisièmement, elle serait dotée d'une mission de contrôle afin de s'assurer que le mécanisme descendant de la planification est atténué par une prise en compte des besoins du territoire. Notre travail en appelle à une réforme du financement de l'accompagnement des personnes handicapées. Les élus qui siègent dans cet hémicycle sont particulièrement informés des inconvénients du cofinancement, par l'agence régionale de santé et le conseil départemental, d'un nombre important de structures chargées de cet accompagnement. pas de réforme efficace de l'accompagnement sans respect scrupuleux d'un principe de financeur unique ! Au-delà de la concurrence des financeurs, c'est le financement des prestations par la personne elle-même qu'il est urgent de repenser et de rationaliser. Le principal instrument de cette réforme à venir est incontestablement la prestation de compensation du handicap, la PCH. Cette dernière doit être profondément simplifiée et devenir le principal appui financier de toutes les dépenses d'accompagnement handicapée, essentiellement les aides humaines et les aides à l'aménagement du logement et du véhicule. Les aides techniques, qui relèvent actuellement de la PCH, alors que leur vocation est essentiellement médicale ou paramédicale, devraient à mon sens être financées par l'assurance maladie. Outre une réduction certaine du reste à charge dont de nombreux usagers doivent encore s'acquitter, cette répartition simple et logique facilitera la vie financière des personnes handicapées qui, perdues entre les divers guichets, caisses et bureaux qui leur sont désignés, multiplient les démarches pour se faire rembourser les frais d'acquisition d'un fauteuil roulant, les frais d'installation de rampes d'accès, les frais de trajet entre domicile et établissement sont, madame la secrétaire d'État, les voeux que formule la commission des affaires sociales à votre intention. Vous avez la responsabilité d'un ministère dont nos concitoyens en situation de handicap ont beaucoup attendu, sans toujours beaucoup recevoir.

Mouiller de me donner, grâce à ce débat et à son excellent rapport, l'occasion de rappeler la pleine convergence du Gouvernement et des sénateurs pour construire une société inclusive, c'est-à-dire une société qui donne pleinement leur place aux personnes en situation de handicap, conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la convention internationale des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Donner pleinement leur place aux personnes handicapées signifie non pas les laisser sans accompagnement,

ne répond pas pleinement à cet objectif. C'est pourquoi le « virage inclusif » de l'offre est au coeur de la feuille de route gouvernementale. La nécessité de cette transformation est apparue dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », engagée à partir du rapport intitulé « Zéro sans solution », élaboré par Denis Piveteau à la demande du Gouvernement. mise en place de dispositifs plus soutenus reste indispensable, notamment pour les personnes présentant les besoins les plus complexes, mais elle ne doit pas constituer la seule réponse possible pour tendre vers ce « zéro sans solution Près de 500 000 places en établissements et services pour personnes handicapées sont aujourd'hui recensées, dont 160 000 pour les enfants et près de 340 000 pour les adultes. Cela représente un budget d'environ 17 milliards d'euros. est de constater que la part des services dans l'ensemble de l'offre, malgré des progrès incontestables, reste insuffisante, en particulier pour les services d'accompagnement des adultes, qui ne représentent que 20 % des réponses. Il nous faut donc changer de cap, faire tomber les murs, raisonner désormais en parcours accompagnés, quatre objectifs prioritaires devant guider notre action : ne pas laisser la personne et ses proches seuls face à l'absence d'un accompagnement faire évoluer l'offre afin qu'elle soit plus inclusive et plus souple ; renforcer la participation des personnes concernées à la mise en place des solutions d'accompagnement ; engager un mouvement de formation pour accompagner ces évolutions et ces professionnels. Cette ambition est soutenue par la mise en oeuvre de la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre médico-sociale, qui permet de mobiliser un financement de 180 millions d'euros afin de proposer des solutions nouvelles et de répondre aux situations les plus complexes. Ces efforts ont été confortés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, avec le triplement des moyens consacrés à la prévention des départs en Belgique et des crédits spécifiques dédiés à la mise en oeuvre de la stratégie pour l'autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux. Ces investissements supplémentaires permettront de développer les nouvelles réponses, très prometteuses, que sont les unités d'enseignement dans les écoles ordinaires, les pôles de compétences et de prestations externalisées, l'habitat inclusif ou l'emploi accompagné. Je souhaite également que l'on puisse diversifier les accompagnements offerts par les établissements et services existants, en proposant des accueils de jour comme de nuit, des accueils temporaires ou séquentiels, ou encore des interventions hors les murs : c'est pour moi essentiel. Cependant, diversifier, développer, transformer ne suffit pas. Nous avons aussi besoin d'assouplir, de gommer ces complexités administratives et financières qui constituent parfois des obstacles majeurs à notre ambition. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite généraliser les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les associations gestionnaires. Cette généralisation devra sans doute être accompagnée, comme vous le proposez, monsieur le sénateur Mouiller, par une clarification des financements, encore trop morcelés, ce qui nuit à la cohérence de notre stratégie. Oui, le chemin vers une société inclusive est encore aventureux, et les territoires doivent être pleinement mobilisés pour organiser cette réponse simplifiée et ajustée à l'ensemble des besoins. Concernant les territoires, il s'agit d'impliquer, comme vous le notez si bien, tous les acteurs susceptibles d'évaluer finement les besoins, d'animer l'évolution de l'offre et de fluidifier les parcours. C'est d'ailleurs tout le sens que j'ai voulu donner à la démarche des « territoires 100 % inclusifs » que j'ai lancée cette année dans le Territoire de Belfort et qui vise à créer cette communauté de regard et d'action entre les acteurs pour accélérer la transformation. J'ai besoin de vous pour concrétiser cette ambition. Le virage inclusif est pris, le mouvement ne s'arrêtera plus. Toutefois, ce virage n'est qu'un des leviers de la transformation profonde à laquelle nous aspirons. des personnes handicapées, la place de nos concitoyens en situation de handicap s'est améliorée, mais le fonctionnement de notre société reste encore trop souvent source d'exclusion et de défiance. C'est la raison

monsieur le sénateur, le Gouvernement s'engage à permettre l'attribution de droits à vie aux personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Cela pourra concerner l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 %, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais aussi l'octroi de la carte mobilité inclusion ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ainsi, les personnes n'auront plus besoin de renouveler, parfois dix fois dans leur vie, les mêmes demandes. Mais ce n'est pas tout : les personnes handicapées majeures sous tutelle vont pouvoir bénéficier d'un droit de vote inaliénable, elles auront le droit de se marier, de se pacser, de divorcer, de se soigner, sans devoir recourir à l'autorisation judiciaire, tout en conservant l'accompagnement par les tuteurs. C'est un progrès considérable qui permettra de reconnaître enfin les personnes handicapées comme des citoyens à part entière, et non plus comme des citoyens à part.

se joue dès le plus jeune âge, une grande concertation nationale vient d'être lancée, conjointement avec Jean-Michel Blanquer, afin d'effectuer le saut qualitatif nécessaire pour consolider l'école inclusive. en matière d'emploi, nous poursuivrons le travail global engagé en faveur du soutien à l'activité des personnes handicapées, conforté par les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et nous rénoverons l'offre de services pour sécuriser les parcours vers et dans l'emploi. En quatrième

et, bien sûr, l'amélioration du repérage des troubles de l'apprentissage et du neurodéveloppement, avec le développement d'un « forfait intervention précoce » dès le 1 janvier 2019. Enfin, le Gouvernement affirme l'ambition très forte de permettre à toutes les personnes d'accéder aux nouvelles technologies pour favoriser leurs communications et leur autonomie. et leur autonomie. Mettre en lien les start-up, les développeurs et les personnes pour concevoir et tester de nouveaux outils constituera ainsi un nouvel enjeu interministériel. Cette société du vivre ensemble s'incarnera également à travers la prochaine Conférence nationale du handicap, qui s'adressera à tous les citoyens et permettra de valoriser les initiatives et les pratiques locales. C'est C'est à cette occasion que nous ouvrirons le chantier très attendu de la prestation du handicap, tant pour les enfants que pour les adultes, notamment pour mieux soutenir la parentalité des personnes en situation de handicap et mieux prendre en charge les besoins de compensation des enfants. Le Gouvernement entend également reconsidérer le statut et la gouvernance des maisons départementales des personnes handicapées pour améliorer le pilotage de l'offre médico-sociale. Parce que cette grande conférence doit être avant tout une dynamique émanant des territoires, des expériences locales, de la vraie vie, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à contribuer à ces échanges, qui nous permettront de construire ensemble ce « droit commun accompagné » et de bâtir une société inclusive qui redonne confiance et dignité. je vous remercie

Quelles garanties avons-nous quant à l'égalité de droits entre citoyens sur le territoire national ? Madame la secrétaire d'État, quels moyens allez-vous donner aux départements pour assumer ce nouveau transfert de compétence ? Quels moyens pour l'inclusion,

dans la cité : les déclarations de principes, c'est bien ; leur concrétisation par des actes politiques, c'est mieux ! Or la réduction du taux de logements neufs accessibles votée par votre majorité lors de l'examen du projet de loi ÉLAN entre en contradiction avec vos orientations proclamées. La politique inclusive recueille l'assentiment majoritaire des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs associations de défense. Ainsi, il est tout à fait logique que les parents soient favorables à l'intégration de leur enfant handicapé en milieu scolaire « ordinaire », avec adaptation aux spécificités du handicap et recours aux auxiliaires de vie scolaire- si tant est que ces derniers puissent être respectés pour leur travail correctement. Mais la réalité, parfois dure à entendre pour les parents, est que tous les enfants handicapés ne peuvent pas suivre une scolarité dans le milieu « ordinaire ». Certains risquent de ne pas trouver leur équilibre en cas d'intégration ratée ou à marche forcée.

Je veux saluer la qualité du travail accompli par les entreprises adaptées et leur rôle essentiel dans l'accompagnement des personnes handicapées. Je rappelle d'ailleurs que, l'année dernière, le Gouvernement avait décidé de baisser les aides destinées à ce secteur, ce qui menaçait, en particulier, 700 emplois dans mon département du Pas-de-Calais. Seule une mobilisation de grande ampleur des acteurs du secteur et des élus a permis le gel de cette mesure, mais l'inquiétude demeure. Je souhaite donc attirer votre attention, madame la secrétaire d'État, sur le fait que si l'avènement d'une société inclusive est évidemment plus que souhaitable, certaines personnes handicapées, plus fragiles, doivent bénéficier d'une intégration dans un milieu qui les protège davantage. Avez-vous conscience du travail mené par les professionnels du secteur protégé, et vous engagez-vous aujourd'hui à ne pas diminuer leurs moyens ? La parole est à Mme la secrétaire

Madame la secrétaire d'État, le 24 mai dernier, alors que je vous faisais part ici même de l'inquiétude des personnes en situation de handicap et de leurs familles, vous m'avez assuré de l'engagement plein et entier du Gouvernement sur le sujet.

pour réaliser les diagnostics et du manque de dispositifs tels que les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, pourtant si nécessaires pour une inclusion réussie dans le milieu scolaire. Par ailleurs, les enfants présentant des troubles « dys

ans après la promulgation de la loi qui devait opérer un changement de regard sur le handicap et mettre fin aux inégalités persistantes dont souffrent les personnes en situation de handicap. Je redis mon inquiétude et j'attends des engagements forts de votre part,

« troubles du neurodéveloppement » a l'avantage d'englober les formes diverses du handicap d'origine neurologique. Elle présente néanmoins le risque d'une assimilation contre-productive contre-productive entre troubles relevant du spectre de l'autisme, troubles de l'apprentissage, troubles de l'attention et troubles liés à la déficience intellectuelle. Les âges de détection des handicaps et les réponses à leur apporter ne sont pas, par définition, les mêmes. L'article 40, en prévoyant une réponse trop globale, manque son objectif. la détermination de l'acteur chargé de l'organisation de ce bilan d'intervention précoce, ensuite, l'article 40 vise les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psychologiques, mais aussi les établissements de santé psychiatrique. Ce dernier point ne laisse pas d'inquiéter les familles, qui peinent encore aujourd'hui à faire reconnaître que le handicap neurologique ne doit pas être traité comme la maladie mentale. L'inquiétude et les craintes liées à l'histoire des pratiques en France, notamment le recours à la psychanalyse, resurgissent : je me réfère à l'excellent rapport élaboré par Valérie Létard en vue de la mise en place du plan

Actuellement, les familles concernées perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, d'un montant de 130 euros mensuels. Cette aide fait l'objet d'un complément déterminé par la commission départementale en fonction du niveau de handicap de l'enfant. Or, comme nous pouvons le constater- et la loi insiste sur ce fait -, il est parfois difficile d'évaluer le degré de handicap chez de jeunes enfants. Certains enfants handicapés ont besoin qu'un aidant

C'est pourquoi les pouvoirs publics doivent leur permettre de conjuguer leur engagement personnel et leur vie professionnelle. Pour ce qui concerne les aidants d'enfants handicapés, en cas de reprise d'activité professionnelle, le montant du complément d'allocation devient dégressif.

Comment le Gouvernement entend-il procéder pour permettre à ces familles, déjà lourdement éprouvées, de bénéficier d'une aide complète tout en conservant une activité professionnelle ? J'ajoute que cette question est indissociable

durant ce quinquennat afin de mener une politique réellement concertée en matière d'accompagnement de la dépendance, quelle qu'elle soit ?

pour la création de places en établissements médico-sociaux entre 2014 et 2018. Pour ce qui concerne plus précisément l'autisme, aucun des deux derniers plans n'a été respecté : 6 752 places devaient être réalisées, seulement 4 465 l'ont été ! La Haute La Haute Autorité de santé estime que 700 000 personnes sont atteintes d'autisme en France, dont 100 000 enfants. Seulement 27 % des enfants sont accueillis dans des structures, dédiées ou pas. Le taux d'accueil tombe à 10 % pour les adultes, ce qui est dramatiquement inférieur aux besoins. Derrière ces chiffres, il y a les attentes et les souffrances des familles. J'ai pris connaissance de la « stratégie nationale pour l'autisme » pour les années 2018-2022 : 1 500 places seront créées, mais il est précisé qu'elles serviront uniquement à l'achèvement du troisième plan Autisme, prévu pour 2017. Les créations de places sont donc figées. Le comité interministériel du handicap assume, pour l'avenir, de « sortir d'une logique de places pour entrer dans une logique de parcours accompagnés », c'est-à-dire de transformer les places existantes au lieu d'en créer de nouvelles. À l'instar de notre rapporteur,

Les parents s'épuisent à garder à leur domicile leurs enfants devenus adultes. Ils mènent un véritable parcours du combattant en multipliant les recherches et en enchaînant les échecs. Ils vivent avec la peur de disparaître avant d'avoir trouvé une solution pérenne, sans laquelle leur enfant serait placé dans un lieu totalement inadéquat, le plus souvent

Théoriquement, la réglementation en vigueur permet une couverture intégrale des dépenses engendrées par le handicap de la personne accompagnée. L'article R. 314-26 du code de l'action sociale et des familles dispose que la dotation médicale de chaque établissement ou service couvre uniquement les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et de laboratoire afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service. Il est complété par la disposition de l'article R. 314-122 du même code en vertu de laquelle tout soin complémentaire délivré à titre libéral à l'extérieur, donc indépendamment du forfait versé à la structure accompagnatrice, est pris en charge maladie de l'ayant droit dans les conditions de droit commun, si ce soin ne peut être assuré par la structure accompagnatrice. Or, dans les faits, des différences d'interprétation de ces dispositions engendrent une hétérogénéité des pratiques des caisses primaires maladie. Certaines s'appuient sur la rédaction de l'article R. 314-26 pour justifier le financement d'interventions de psychologues, d'ergothérapeutes ou de psychométriciens, d'autres pour refuser leur prise en charge,

À titre préliminaire, je tiens à saluer la qualité des travaux menés par mon collègue Philippe Mouiller. Je m'associe pleinement aux préconisations formulées par son groupe de travail. Madame la secrétaire d'État, ma question portera sur l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes et, plus particulièrement, sur les démarches administratives Beaucoup de formulaires à remplir sont actuellement disponibles en version papier. Toutefois, l'heure est à la dématérialisation des procédures, qui, j'en suis sûre, s'étendra à l'ensemble de ces personnes.

39 % des personnes âgées de soixante-dix ans et plus estiment que les équipements comme les ordinateurs, les tablettes et les smartphones sont « plutôt difficiles » ou « très difficiles » à utiliser. Diverses initiatives locales sont prises pour traiter cette problématique. À titre d'exemple, un bus numérique a été mis en place dans la région Centre-Val-de-Loire.

d'autonomie. Cette instance a été mise en place par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Elle constitue un levier d'accompagnement des actions individuelles ou collectives destinées aux personnes âgées de soixante ans et plus.

En dix ans, le nombre d'élèves handicapés a triplé dans les établissements relevant de l'éducation nationale : il est passé de 100 000 en 2006 à 320 000 en 2017. Cette augmentation est l'une des conséquences de la loi du 11 février 2005, qui a rendu obligatoire l'inclusion scolaire des enfants porteurs de handicap. Les professionnels qui accompagnent ces élèves handicapés jouent un rôle fondamental pour leur intégration dans le système scolaire. Toutefois, le statut de ces « héros du quotidien » n'est pas à la hauteur de la tâche qui est la leur.

des élèves en situation de handicap, présentée par notre collègue député Aurélien Pradié, en est la meilleure illustration. La rémunération ne doit pas être la principale motivation des personnes exerçant ce métier si particulier, nous en convenons. Mais, vous en conviendrez également, madame la secrétaire d'État, la rémunération ne doit pas être le principal frein à l'attractivité de cette profession.

et outiller les enseignants ; c'est l'objet de la plateforme numérique qui sera développée au cours de cette année. Elle permettra une adaptation pédagogique selon les troubles, selon les retards d'apprentissage, quel que soit le type de handicap.

l'objectif étant de faciliter l'insertion, d'ancrer la notion de parcours dans l'accompagnement médico-social et de mettre en place des passerelles entre milieux ordinaire, adapté et protégé. Les MDPH constituent, selon moi, des acteurs départementaux incontournables en raison de leur connaissance fine du territoire, qui les met en mesure de produire un véritable recensement qualitatif des besoins de la population, étape fondamentale en vue de la réalisation d'un diagnostic territorialisé et prospectif.

sont bien intégrés dans le paysage départemental depuis les années 2000. Ces guichets uniques d'information et d'accompagnement social dédiés aux personnes âgées, répartis au plus près des territoires, sont capables de rendre un véritable service de proximité.

conforme à la proposition du rapporteur visant à rendre aux conseils départementaux un rôle décisif en matière de planification de l'offre médico-sociale. Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous donner votre sentiment sur cette proposition ? La parole est à Mme la secrétaire d'État.

En théorie, depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises ont l'obligation de compter 6 % de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. En pratique, ce taux n'est que de 3,5 %, les entreprises préférant payer une contribution plutôt que d'embaucher

Il faut favoriser la rencontre entre l'entreprise et la personne handicapée, qui constitue bien souvent un choc positif pour l'entreprise, crée de la solidarité et permet d'accompagner les personnes handicapées vers l'indépendance. Il nous faut donc agir pour favoriser l'insertion dans le milieu professionnel ordinaire, même si les entreprises du secteur adapté font un travail remarquable, comme je peux le constater dans mon département de la Mayenne. Le rapport de notre collègue Philippe Mouiller met en exergue plusieurs difficultés qui expliquent la réticence des entreprises du milieu dit « ordinaire » à embaucher des personnes handicapées. Par exemple, l'orientation et l'insertion professionnelle de ces dernières sont des missions de Pôle emploi, de Cap emploi et des missions locales,

Il constitue un levier pour la transformation de l'offre de services en faveur des personnes handicapées, qui doit s'inscrire dans une réflexion globale. Cette réflexion nécessite une anticipation suffisante

plus loin, que « l'intention de départ, consistant à partir des besoins des personnes pour construire la nouvelle tarification, est parfaitement louable, mais le chemin que prend la réforme, loin de faire " tomber les murs " autour de la personne, ne paraît en fait que modifier leur agencement. L'ambition première de la réforme risque de se voir passablement émoussée par un tropisme [ ...] consistant à voir dans la réforme tarifaire l'outil principal de restructuration de l'offre.

Au vu des préconisations contenues dans le rapport sénatorial, le calendrier de la réforme ne doit-il pas être revu, afin de se donner le temps d'analyser les incidences de ce nouveau modèle tarifaire et d'associer les acteurs à la définition des dispositifs transitoires ?

pour établir enfin un lien direct entre les modalités de l'accompagnement proposé, le public accueilli et le niveau de budget alloué. Notre intérêt collectif est bien de mettre fin à cette grande dispersion des coûts promouvoir un nouveau modèle de financement. Cette orientation a été confortée dans le cadre du lancement de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ». Dans ce contexte, le projet SERAFIN-PH doit permettre d'apporter toutes les souplesses nécessaires pour ajuster le financement des établissements à la complexité de certaines situations individuelles. Je voudrais vous rassurer sur la méthode de travail qui a été suivie. Ce projet est un chantier de long terme, qui a fait toute sa place à la concertation et à la coconstruction avec les différents acteurs, en particulier dans le cadre du groupe technique national. Il a été planifié pour se dérouler en trois phases et s'étendra sur plusieurs années. première phase, engagée en 2014, a pour objet de concevoir les outils qui permettent de rénover le modèle d'allocations. Il s'agit d'élaborer concrètement les nomenclatures de besoins et de prestations, qui ont été validées en 2016, et de mener des enquêtes et des études nationales de coûts. Deux enquêtes ont ainsi été réalisées, en 2016 et en 2017, et la première étude étude nationale sera engagée cette année. Les phases 2 et 3 viseront à étudier et à définir de nouvelles modalités de tarification, puis à les déployer. À ce stade, aucun choix n'a donc été prédéfini ni arrêté, et le projet ne vise en aucun cas à remettre en cause la qualité des accompagnements des personnes.

et les membres du groupe de travail pour cet excellent rapport d'information. Aujourd'hui, le contrôle par les pouvoirs publics de l'offre médico-sociale à destination des personnes handicapées relève de trois échelons territoriaux, dont les rôles sont parfois difficiles à distinguer pour les utilisateurs. En premier lieu, l'État élabore un schéma pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes dont les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau. La planification nationale prend la forme de grands plans pluriannuels, généralement annoncés par le chef de l'État dans le cadre triennal de la conférence nationale du handicap. le représentant de l'État dans la région, appuyé par les services de l'ARS, établit les schémas régionaux de l'offre médico-sociale relatifs aux établissements et services accueillant des personnes handicapées.

En effet, détenteur d'une compétence générale en matière sociale depuis les lois de décentralisation, compétence qui a été confirmée par la loi du 27 janvier 2014, le département aurait dû naturellement prétendre à la coordination et à l'organisation de l'offre médico-sociale sur son territoire.

leurs attentes. Le schéma de l'offre médico-sociale du département est réellement complémentaire des schémas régionaux en matière de planification de l'offre. N'oublions pas que le département reste le premier à connaître les besoins exprimés et doit, à ce titre, être à l'origine de la décision de création de l'offre.

vous remercie, madame la secrétaire d'État, des réponses que vous avez apportées à nos collègues et de l'accueil que vous faites régulièrement au travail parlementaire. J'aime à souligner que sa publicité n'est souvent pas à la mesure de son utilité

dont l'application peut parfois nuire gravement à la pertinence des soins prodigués. Or j'ai souvenir que, au moment du lancement de sa réflexion, le groupe de travail sénatorial sur le financement de l'accompagnement du handicap s'est longuement interrogé sur l'avenir d'une réforme tarifaire des établissements et services médico-sociaux accueillant les personnes handicapées engagée par le Gouvernement en 2014, mais dont l'aboutissement n'est toujours pas connu avec certitude : je veux parler de la réforme SERAFIN-PH. Bien qu'elle soit éclipsée par l'actualité,

le rappelle, d'extraire l'attribution des crédits versés par le financeur d'une stricte logique de reconduction des dotations historiques et d'enfin faire correspondre les besoins réels des personnes handicapées admises dans des structures d'accompagnement et l'allocation de l'argent public qui finance ces structures. Je note avec inquiétude que cette réforme, que tout le monde s'accordait à dire bien engagée, montre quelques signes d'essoufflement et prend une tournure différente de celle qui avait été initialement annoncée. Les conclusions de notre rapporteur ont effet mis en lumière que les besoins en matière de santé somatique et psychique des personnes handicapées faisaient certes l'objet d'un repérage et d'une nomenclature affinée, mais que leurs besoins socio-éducatifs beaucoup moins précisément retracés. Or, madame la secrétaire d'État, la tarification à l'acte médico-social- si vous me permettez d'utiliser ce raccourci -n'a justement rien à voir avec la tarification à l'acte médical, dont il semble pourtant qu'elle se rapproche dangereusement. C'est tout à fait inexact ! Vous aurez l'occasion de revenir sur le sujet ! C'est tout l'enjeu de la société inclusive, dont il n'a cessé d'être question, que de démédicaliser l'accompagnement des personnes handicapées et de revaloriser fortement sa dimension humaine et sociale. Je conviens que cette tâche est particulièrement ardue. Quantifier les besoins en santé a toujours été plus aisé